Les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont d'ailleurs émis des propositions fortes sur le sujet, en rappelant que la publicité a des effets très sensibles sur la création de besoins et la consommation. Ils ont ainsi suggéré de fixer une trajectoire d'interdiction des publicités en faveur des produits ou services ayant un impact environnemental excessif et de mettre dès à présent en place des interdictions plus ciblées, par exemple sur les véhicules frappés d'un malus écologique.

de professionnels, lesquels sont censés prendre, depuis des années, leur part de responsabilité en matière environnementale et climatique ... Or la publicité continue de promouvoir un modèle privilégiant la surconsommation alors que la transition écologique suppose un monde plus sobre, soucieux des limites planétaires et de l'empreinte écologique des activités humaines.

réellement pour promouvoir des produits, des services et des imaginaires compatibles avec la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. Le groupe socialiste défendra un certain nombre de propositions relevant d'une stratégie de bon sens pour une

Parce que la publicité progresse partout et modèle les espaces urbains, nous voulons donner aux élus locaux les moyens de réinvestir les centres-villes et de réguler

Demilly. L'article 4 vise à interdire toute publicité pour les énergies fossiles. Or les secteurs concernés par l'interdiction, qui ont déjà été fortement touchés par la crise sanitaire, doivent réaliser d'importants investissements technologiques pour s'adapter aux enjeux écologiques. Leur imposer une restriction de communication durant une crise sanitaire et économique comme celle que nous vivons n'est pas très opportun, alors même que nombre d'entre eux s'engagent fortement dans la transition écologique. Je pense notamment à une grande entreprise française comptant 100 000 collaborateurs répartis dans 130 pays.

Le centre de recherches en question lui attribue la note de 97 sur 100 et la positionne sur la troisième marche mondiale parmi les quatre secteurs étudiés. La mesure prônée à l'article 4 privera de recettes les médias audiovisuels et radiophoniques, ainsi que la presse écrite, mais également les collectivités locales, qui perdront les recettes issues de la taxe locale sur la publicité extérieure.

la réalité de l'exposition publicitaire des citoyens est extrêmement difficile à évaluer, mais elle fait l'objet de quelques estimations. Dans un ouvrage de 2007, Arnaud Pêtre estime que les Français sont exposés à 15 000 commerciaux par jour et par personne.

Les modalités d'application sont renvoyées à un décret destiné à définir plus finement les catégories de biens concernés, mais nous souhaitons d'ores et déjà inclure au dispositif les véhicules, certaines liaisons aériennes, ainsi que certains produits électroménagers. Cette nouvelle rédaction renforcerait considérablement l'article et permettrait d'amorcer réellement les changements en matière de publicité

Le Conseil d'État et d'autres organismes, comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE), ont souligné la faible portée de l'article 4 sur l'encadrement de la publicité. Les mesures proposées ne permettent pas de considérer le projet de loi comme adapté et proportionné à l'objectif visé : diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession devra s'engager- nous y reviendrons -, il nous paraît nécessaire de fixer quelques règles essentielles qui devraient s'appliquer à toutes les publicités. Cet amendement vise ainsi à acter un principe : toute publicité, quel qu'en soit le support, faisant la promotion de biens ou de services respecter les principes et les objectifs de développement durable adoptés par l'assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. Cela nous semble être le préalable de toute régulation de la publicité. libellé : La parole est à M. Stéphane Demilly. D'après l'avis du Conseil d'État sur l'article 4, l'expression très générale utilisée dans le projet de loi ne permet pas de savoir si l'interdiction vise uniquement des publicités directes pour une source d'énergie n'incluant pas de référence à un produit utilisant l'énergie ou si elle concerne aussi des publicités se référant à la fois à une énergie et à un produit consommateur d'énergie. Le présent amendement de repli vise donc à réécrire l'alinéa 5 pour préciser que l'interdiction porte spécifiquement sur la publicité directe en faveur des énergies fossiles.

passer par une incorporation progressive d'énergies renouvelables dans un constitué d'énergies fossiles. Cet amendement de repli vise à préciser le texte pour que le décret pris en Conseil d'État garantisse bien la possibilité, pour ces énergies renouvelables incorporées ultérieurement à des énergies fossiles, de faire l'objet de publicité.

Le gaz naturel émet trois fois moins de CO2 par kilowattheure d'électricité produite que le charbon, à telle enseigne, d'ailleurs, que le remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz est le principal facteur d'explication de la baisse des émissions de CO2 par habitant intervenue dans certains pays.

En effet, les biocarburants sont des carburants de substitution obtenus à partir de la biomasse, qu'il s'agisse de matière première d'origine végétale, animale ou issue de déchets. Leur contenu biogénique est donc, par définition, de 100 %. Ils sont généralement incorporés dans les carburants d'origine fossile ; nous le savons tous. l'objectif de l'article est bien d'exclure les carburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.

En effet, un large consensus émerge autour de l'idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs, en mobilisant un imaginaire contradictoire avec les discours raisonnés d'utilisation sobre et économe des ressources. Selon Bernard Stiegler, le marketing détruit tous les outils du savoir. La raison est simple : le marketing but de prendre le pouvoir sur le psychisme de l'individu, afin de l'amener à un comportement pulsionnel. Cette captation est évidemment destructrice. On canalise le désir vers des moyens industriels et la consommation à outrance. Pour cette raison, il nous semble urgent de contrôler la publicité et les messages régressifs

Là encore, notre amendement est en cohérence avec d'autres propositions que nous défendrons plus loin. Notre groupe souhaite qu'il soit mis un terme à la vente des véhicules neufs les plus émetteurs de gaz à effet de serre d'ici à 2025 et à celle des véhicules thermiques en 2030,

et plus difficiles à manoeuvrer, sont également extrêmement polluants à la fabrication. Même si celle-ci a souvent lieu en dehors de nos frontières, sous d'autres cieux, il nous appartient de remédier des solutions locales à un problème global a toujours été notre. Je profite également de cette parenthèse pour réaffirmer avec force que le tout-électrique ne saurait être une solution viable. La véritable solution, c'est la réduction des trajets réalisés par des véhicules individuels, en favorisant le report modal par tous les moyens, en complément des mobilités actives. Surtout, l'article 4 tel qu'il résulte des travaux de la commission prévoit l'interdiction de la publicité pour les véhicules polluants en 2028. Un tel délai nous paraît inutilement long au vu de l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés. C'est aujourd'hui qu'il faut agir de toutes nos forces pour ne pas aller

M. Joël Bigot. La neutralité carbone à l'horizon de 2050 suppose la disparition ou la très forte limitation de certains produits ou services particulièrement polluants. Le présent amendement vise à acter l'interdiction de toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion de biens dont la disparition est programmée. Nous proposons que le délai entre la date d'interdiction de la publicité et celle du produit précédant l'échéance soit fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit. On ne peut pas maintenir la publicité pour des produits dont la vente va être interdite. Ce ne serait ni cohérent ni lisible pour nos concitoyens.

Atteindre les objectifs que la France s'est fixés, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone, implique de fixer des trajectoires pour l'ensemble des acteurs économiques. acteurs du secteur de la publicité doivent s'inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence. Aussi, au travers de proposons d'interdire la publicité pour les biens ayant un impact négatif sur l'environnement, et ce à compter du 1 janvier 2024.

parole est à M. Joël Bigot. Les véhicules les plus polluants font l'objet d'une étape intermédiaire dans le processus d'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques à l'horizon de 2030. Considérant que la durée moyenne de détention d'une voiture est de huit ans ou neuf ans et que l'achat d'une voiture neuve est un investissement important pour les ménages, la transparence et la bonne information du consommateur impliquent que ces véhicules ne fassent plus l'objet de campagnes de publicité dans des délais raisonnables. Aussi, au travers de cet amendement, nous proposons une interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants à compter du 1 janvier 2023. La date du 1 janvier 2028, retenue par la commission, nous paraît bien trop tardive eu égard aux enjeux pour les ménages. Varaillas. Nous avons soutenu en commission l'adoption de l'amendement, important, visant à interdire la publicité sur les véhicules les plus polluants, reprenant ainsi une

Les SUV, du fait de leur poids et de la puissance de leur moteur thermique, émettent environ 25 % de plus de CO2 que les voitures de taille moyenne. Ils sont par ailleurs plus accidentogènes.

Par ailleurs, les publicités pour des SUV occupent chaque jour l'équivalent de dix-huit pages dans la presse et trois heures cinquante à la télévision, représentant une somme de 1,8 milliard d'euros. Grâce à ce marketing intensif dans l'hexagone, les ventes de SUV ont été multipliées par sept en dix ans et représentent aujourd'hui près de 40 % des ventes de voitures neuves. Cette pollution doit cesser rapidement, et le message doit être entendu par les industriels. Nous souhaitons donc aller plus loin, en interdisant ce type de publicités dès 2024.

les conséquences de la production textile à base de microfibres plastiques. Sans une telle information, les procédés de fabrication et leurs conséquences sur l'environnement restent inconnus du consommateur. Je suis déjà intervenue sur le sujet hier. Je rappelle que la croissance de la consommation textile- 40 % en plus ces quinze dernières -est

en haut du Pic du Midi, dans les sédiments, dans l'air et dans toute la colonne d'eau des rivières, des océans et des mers. Les microfibres sont « relarguées » en continu, tout au long de leur cycle de vie,

du lavage en machine : de 700 000 à 17 millions de microfibres, suivant les tissus. Les microfibres ne se décomposent pas dans l'environnement. Elles vont rester des centaines d'années.

de maladies. On a déjà constaté que les dinoflagellés chez les huîtres pourraient provenir de cette pollution plastique. Les microfibres « relarguent » également tous les additifs qu'elles contiennent les colorants, les retardateurs de flamme. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'un sujet de santé publique, mais aussi de biodiversité. Ces microfibres ont un effet délétère sur la microfaune marine et des sols, notamment sur les vers de terre, qui- vous le savez -sont absolument indispensables. Il y a donc urgence à limiter le flux massif d'arrivées de ces microfibres Nous proposons donc que toute publicité en faveur de la commercialisation d'un bien contenant un textile à base de microfibres plastiques soit assortie d'un message précisant que la production, l'utilisation et l'usage de ce bien « relarguent » des microfibres dans l'environnement.

L'amendement n° 1397 me semble porter une atteinte forte et disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Par ailleurs, au-delà des interdictions de publicité ciblées que nous avons prévues- énergies fossiles, véhicules polluants -, la commission a validé, renforcé et consolidé la logique d'autorégulation, sous l'égide du CSA,

L'amendement n° 74 rectifié soulève des difficultés juridiques, qui avaient été levées lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale pour tenir compte des remarques sévères du Conseil d'État sur cet article. Viser la Viser la publicité directe en faveur des énergies fossiles est trop imprécis par rapport à la commercialisation, la promotion ou la vente de ces énergies. Je propose donc d'en rester à la rédaction juridiquement

L'amendement n° 2028 rectifié tend à revenir sur la position de la commission et le travail que nous avons effectué avec Daniel Gremillet pour prévoir des exceptions relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants.

L'amendement n° 346 me paraît en décalage avec les capacités de transformation de notre industrie automobile. Il comporte également une interdiction très large, qui porterait atteinte au financement de nos médias.

de mentions spécifiques pour les produits textiles à base de microfibres plastiques. Je suis réservée sur l'ajout de nouvelles mentions dans les publicités. Il en existe déjà des centaines et toutes ne sont pas bien positionnées, du fait de la difficulté de les inclure dans les supports. La pollution

en renforçant la mise en avant des produits et des comportements ayant moins d'impact sur l'environnement. Une vraie dynamique s'est d'ailleurs enclenchée, du côté des annonceurs comme des agences de médias. En complément des dispositions qui, au sein de l'article 4, vont rendre obligatoire l'affichage

rectifié vise à supprimer la précision selon laquelle le décret en Conseil d'État fixe les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. Nous

Le Gouvernement rappelle que l'article 4 a vocation à interdire la publicité en faveur d'une liste d'énergies fossiles. Par définition, les énergies renouvelables sont exclues de cette interdiction. Se pose dès lors la question des mix énergétiques incluant à la fois des énergies fossiles et renouvelables en proportions très variables, pour lesquels le Gouvernement a choisi de se laisser une marge de manoeuvre. Le décret qui fixera la liste des énergies fossiles précisera donc également les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées,

n° 1402 sur la publicité pour les véhicules les plus polluants, j'ai déjà expliqué pourquoi j'étais défavorable à ce genre de dispositions.

par le présent article avec l'article 131-38 du code pénal, qui prévoit que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Ce faisant, il tend à aligner les sanctions prévues au présent article sur celles prévues par la loi dite Évin pour les dispositions comparables d'interdiction de publicités concernant le tabac et ses produits dérivés.

Si l'on suit la logique de la commission, qui a ajouté des sanctions pour défaut de déclaration, celles-ci ne pourraient pas être mises en oeuvre sur la base d'une liste éditée par un acteur privé. En outre, il est utile d'envisager cette déclaration de matière concomitante à la mise à disposition du public des codes de bonne conduite prévus à l'article 5. Or ces codes s'adressent à la fois aux entreprises des filières de communication et médias, mais aussi aux annonceurs qui n'interagissent pas directement avec l'ARPP. Dans un objectif de lisibilité, il est donc souhaitable que la liste des entreprises qui souscrivent et ne souscrivent pas à un code de bonne conduite et les engagements eux-mêmes soient disponibles sur un même espace. Pour ces différentes raisons, je vous propose d'adopter cet amendement, ce qui rendra le dispositif de déclaration des entreprises plus lisible et plus efficace.

L'amendement revient également sur la logique d'autorégulation portée par le projet de loi sur le volet publicité, au-delà des interdictions ciblées sur les énergies fossiles ou les véhicules très polluants. Je ne partage pas cet objectif. Certes, le présent article revient à confier des prérogatives importantes aux autorités de régulation du secteur et à l'ARPP en particulier, mais il me semble nécessaire que ces acteurs s'engagent clairement dans une démarche positive pour l'environnement.

Les mentions obligatoires dans les publicités sont nombreuses, ce qui peut les rendre contre-productives et nuire à leur bonne intelligibilité par les consommateurs. Aussi est-il nécessaire de réserver cet outil d'information des consommateurs à des messages spécifiques visant à remédier à un déficit d'information pour un produit ou service précis, dont les caractéristiques particulières justifient de limiter la liberté du commerce. En l'occurrence, une mention obligatoire très générale sur les risques de la consommation excessive ne permet pas de viser la consommation d'un produit ou service en particulier, dont il serait avéré qu'il nuit à l'environnement. cette mention serait même ajoutée aux publicités pour des produits de faible empreinte carbone ou contribuant à la sauvegarde de l'environnement. S'il convient d'encourager une consommation responsable et écologique, sur laquelle doit se fonder la relance de l'économie, il serait contre-productif de stigmatiser la consommation en tant que telle. La parole

de rendre obligatoire l'affichage environnemental sur les produits comme sur les publicités. Ce sera un affichage simple, lisible, qui se verra du premier coup d'oeil et qui assurera du coup un très haut niveau de transparence pour les consommateurs, lesquels seront ainsi en mesure de faire des choix

l'offre d'un concessionnaire local tenant en deux mots : malus offert ! Ainsi, ce concessionnaire proposait à ses clients de prendre à sa charge le malus automobile dans une sorte de remise promotionnelle. À chaque renforcement des barèmes du malus écologique, des concessionnaires mettent en place des opérations de déstockage préventif de véhicules neufs qui tomberont sous le coup de ces nouveaux barèmes. La loi est la même pour tous et il n'est pas concevable que des annonceurs proposent à leurs clients d'en annuler les effets. Ce qui serait scandaleux dans tout autre domaine devient inacceptable dès lors qu'il s'agit du réchauffement climatique.

que certains annonceurs et agences ne s'en rendent pas compte ! L'adoption de cet amendement permettrait de créer une base légale pour interdire ces pratiques ; c'est donc tout naturellement que j'émets un avis favorable.

article, tel qu'il est rédigé, pourrait être considéré comme non conforme au droit de l'Union européenne, qui interdit de modifier la liste des caractéristiques essentielles d'un bien ou d'un service à partir desquelles une allégation ou une indication fausse ou de nature à induire en erreur peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. En revanche, il est tout à fait possible de rattacher le délit d'écoblanchiment à une catégorie de pratiques commerciales trompeuses consacrée par le droit européen. Par cet amendement rédactionnel, nous proposons de modifier à cette fin le deuxième alinéa de l'article 4 A. Le sous-amendement

elle maintient l'objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse en matière environnementale. L'article L. 132-4 du code de la consommation précise déjà que, en cas de condamnation pour pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs de condamnation. Cette peine complémentaire s'applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse. Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 4 B sont donc redondantes et peuvent, en conséquence, être supprimées. Quel

Le blanchiment écologique se voit qualifié de pratique commerciale trompeuse ; il sera donc sanctionné comme tel. Il devra par ailleurs être interdit d'affirmer à tort dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone. L'écoblanchiment, parfois appelé, sème en effet la confusion dans l'esprit du consommateur, qui ne peut plus distinguer les entreprises, produits et services vertueux sur le plan environnemental de ceux qui n'en ont

Les résultats ont été publiés en début d'année : il en ressort que, dans plus de la moitié des cas, les allégations environnementales des plateformes ainsi visées n'étaient pas étayées par des preuves dans 42 % des cas, l'allégation pouvait être fausse ou fallacieuse et constituer de ce fait une pratique commerciale déloyale en vertu de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. L'objectif de cet amendement est de renforcer le dispositif de lutte contre l'écoblanchiment, en rendant possible l'affichage d'une sanction

? Effectivement, une telle possibilité est déjà prévue. En outre, l'amendement limite la liberté de choix du tribunal, en l'obligeant à choisir la diffusion sur le site internet et la diffusion sur les futures publicités de produits de même catégorie pendant une durée de trente jours, ce qui porte atteinte au principe d'individualisation des peines, qui est de valeur constitutionnelle. Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement

Aller au-delà et interdire purement et simplement la communication sur la neutralité carbone d'une entreprise en considérant que c'est toujours à tort qu'une entreprise communique sur le sujet, puisqu'une telle mention n'est pertinente qu'à l'échelle d'un pays,

citoyens-consommateurs, entreprises, associations, pouvoirs publics -est concerné par cette mutation de notre économie et il ne faut décourager personne d'entreprendre et d'investir dans des stratégies qui visent à réduire l'impact carbone. De nombreuses entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, se sont déjà engagées dans des démarches vertueuses en vue de la préservation des ressources et de l'environnement, tout en assurant une grande qualité des produits destinés à nos concitoyens. Les entreprises sont profondément engagées pour compenser et réduire les émissions de leurs productions elles tendent à être globalement neutres en carbone. Elles doivent pouvoir en faire état dans leurs communications afin d'informer au mieux le consommateur sur les efforts et les actions qu'elles mènent. De plus, les acteurs économiques sont déjà contraints par la législation, en ce sens qu'une allégation fausse ou non prouvée ne peut être utilisée. L'article ainsi rédigé fera peser des contraintes fortes sur les TPE et les PME, pour lesquelles une certification neutralité carbone selon des critères élargis serait extrêmement coûteuse.

Nous avons jugé opportun d'encadrer l'utilisation de la notion de neutralité carbone, qui n'a aucune légitimité scientifique à une autre échelle que nationale ou supranationale et qui peut par ailleurs induire le consommateur en erreur,

j'adhère complètement à cette position. Il faut encourager les démarches vertueuses des entreprises qui souhaitent financer des projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cette raison que le ministère de la transition écologique a mis en place et soutient fortement le développement du label Bas-carbone- c'est un exemple. Il faut que les entreprises puissent faire la promotion de leurs actions et de leur contribution positive à l'action climatique. Néanmoins, appliquer la notion de neutralité carbone à un produit ou service ne trouve pas de justification technique. Comme le mentionnait Mme la rapporteure, une note de l'Ademe parue le 1 avril 2021 indique que la neutralité carbone peut être envisagée à l'échelle nationale ou internationale, mais pas à partir d'un seul produit. Le périmètre d'un produit ou d'un service est trop restreint pour que cette notion ait un sens. Le Gouvernement est très attaché à lutter contre le. La neutralité carbone devient pour de nombreux produits un argument marketing, qui peut tromper le consommateur en lui laissant croire que le produit n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Toutefois, je considère aussi qu'il faut encourager les entreprises à compenser leurs émissions résiduelles et à le faire en toute transparence. C'est pourquoi le Gouvernement proposera un amendement qui, à défaut d'utiliser l'expression « neutralité carbone », permet de substituer intégralement compensé en carbone ». L'utilisation de cette expression est factuellement exacte et nous proposons de l'assortir d'une mise à disposition du public des informations relatives à la manière dont est réalisée la compensation. Cette amélioration de la transparence permettra aux entreprises les plus vertueuses de sortir du lot. Dans la mesure où il nous paraît essentiel d'empêcher toute tromperie du consommateur, je vous suggère de retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement que nous examinerons dans quelques instants. Madame Joseph,

ne dirai que quelques mots : interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir

Demilly. Je suis comme mes collègues Jean-Pierre Grand et Else Joseph dans l'attente des bonnes nouvelles qui devraient tomber dans quelques minutes. Je ne comprends pas cet article, qui introduit l'interdiction générale pour les opérateurs de mentionner la neutralité carbone des produits ou des services sur les emballages ou dans les publicités. C'est une interdiction qui apparaît trop restrictive, car, aujourd'hui, de nombreux acteurs du secteur sont fortement engagés dans une démarche de neutralité carbone certifiée par des tiers extérieurs indépendants, sur la base de référentiels reconnus au niveau européen ou international. Je pense notamment aux certifications ISO. Pour les opérateurs qui s'engagent, cette démarche de neutralité carbone signifie non pas uniquement la compensation des émissions de gaz à effet de serre et l'achat de crédits carbone, mais également l'évitement et la réduction des émissions sur sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Cet engagement est vérifiable d'une manière indépendante et ne peut pas être considéré comme du, me semble-t-il. Une interdiction trop générale constituerait un empêchement pour les entreprises qui se mobilisent et investissent de façon conforme aux engagements pris par la France, l'Union européenne et d'autres pays dans le monde. Cet amendement vise donc à permettre aux opérateurs certifiés de pouvoir continuer à informer le consommateur sur leur engagement pour la neutralité carbone, lorsque celui-ci est prouvé, dans un cadre reconnu, respecté et transparent. On demande aux entreprises d'être vertueuses, mais surtout de ne pas le dire. Ce n'est pas cohérent

Les raisons sont très précises. Avec les autres amendements, il est en fait proposé d'encadrer l'utilisation de la notion de neutralité carbone pour un produit ou un service au lieu de l'interdire, afin que les entreprises puissent communiquer sur leurs actions de compensation. Je rappelle la note de l'Ademe, qui spécifie bien que la neutralité carbone peut être envisagée à l'échelle nationale ou internationale, mais pas à partir d'un seul produit précisément. Attachée à un produit ou un service, cette notion est donc trompeuse pour le consommateur. On comprend bien la logique des amendements et la référence qui est faite aux travaux en cours pour l'élaboration d'une norme ISO

alléguer la neutralité carbone d'un produit ou d'un service revient à mettre en avant une démarche de compensation, étant précisé que c'est la dernière étape de la séquence « éviter, réduire, compenser ». « Compenser » ne peut évidemment en aucun cas se substituer à « éviter et réduire La compensation peut être réalisée de manière plus ou moins vertueuse, à des coûts très différents. Par exemple, 1,5 euro la tonne de CO2 pour des projets d'énergies renouvelables dans les pays en développement, pour lesquels l'additionnalité est assez questionnable, et jusqu'à 10 à 15 euros la tonne de CO2 pour des projets de reforestation qui sont vraiment vertueux. Dans les deux cas, on parle de compensation, et vous voyez bien que l'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. En l'état actuel des travaux sur la norme ISO 14068, les projets les moins vertueux de compensation carbone seraient toujours éligibles pour démontrer la neutralité carbone d'un produit ou d'un service. Dans ces conditions, les garanties de transparence pour les consommateurs ne sont pas réunies. Toutefois, il ne s'agit pas de décourager les entreprises qui s'engagent sur la neutralité carbone de leurs activités, ni celles qui souhaitent développer plus de compensation carbone pour leurs émissions résiduelles. C'est pourquoi le Gouvernement propose cet amendement, cet amendement, qui permet de dissocier une communication sur la neutralité carbone d'un produit ou d'un service d'une communication sur un engagement à la neutralité carbone d'une entreprise. Nous suggérons de communiquer sur des produits intégralement compensés en carbone, tout en rendant publique la manière dont la compensation est réalisée, ce qui permet précisément d'identifier

carbone, s'appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus aux niveaux français, européen et international. Cet amendement devrait pouvoir satisfaire les souhaits formulés par les uns et les autres. est l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune ? Il semble indispensable de mieux encadrer l'utilisation de la notion de neutralité carbone, trop souvent source de confusion pour le consommateur, et ne correspondant pas,

J'ai été, à l'époque, rapporteur des Grenelle de l'environnement I et II. Cela a duré longtemps, beaucoup plus longtemps que ce texte va nous occuper. En particulier, j'avais proposé que les bouteilles en verre soient consignées.

l'affichage, à tort, de cette neutralité carbone article par article, produit par produit. Je trouve que cela revient quand même un peu à prendre les consommateurs pour des imbéciles. Une entreprise peut avoir une stratégie

ayez une démarche globale sur une stratégie d'entreprise, mais, en revanche, arrêtez de prendre les consommateurs pour des idiots en affichant qu'un produit est neutre en carbone.

intéressants, avec du développement et des flux financiers dont nous avons besoin, y compris à l'échelle mondiale, pour la reconquête de la biodiversité et la restauration des puits de carbone. Mais tout va se jouer sur les standards.

qui est discutable et difficile à établir, ou s'agit-il, au contraire, d'encourager les entreprises qui ont la volonté de décarboner des process, qui, aujourd'hui, ne le sont pas

puissent valoriser leurs efforts de décarbonation des process, même s'ils sont tant s'en faut neutres.

Il me paraît donc beaucoup plus important d'encourager les grandes entreprises qui produisent de l'hydrogène à en produire du décarboné, même si l'on sait qu'atteindre cet objectif prendra sans doute une dizaine d'années, sans aucune perspective de neutralité à très court terme. Cependant, il vaut mieux réduire quelque chose d'important et de gênant que de sanctifier des situations très particulières, où le créateur d'un service ou d'un produit aura le privilège, pour des raisons techniques, de ne pas émettre de CO2. Laissons aux entreprises

plus efficaces, plus claires pour nos concitoyens. Nous avons aussi développé le label Bas-carbone, qui est un outil apprécié et efficace, y compris pour nos agriculteurs, d'ailleurs, pour travailler sur les questions de compensation. Ce travail en cours

à nos concitoyens que certaines entreprises vont dans la bonne direction, alors que, clairement, elles utilisent la compensation comme un outil marketing, et certainement pas comme un outil pour la planète. La parole est

; si tel n'est pas le cas, il peut être poursuivi. Cela étant dit, quand on a regardé de près les amendements proposés à la fois par Mme la rapporteure et par vous-même, madame la ministre,

de freiner des entreprises qui souhaitent aller dans le bon sens pour afficher une neutralité carbone. Il y a évidemment la position du Gouvernement, à l'autre extrémité, avec une démarche beaucoup plus compliquée et qui sera beaucoup plus contraignante pour les entreprises. Il y a une autre position, plus modérée, médiane, qui vise à accorder une labellisation de neutralité en carbone, sous

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez. Notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a interdit, à raison, la mention relative au caractère gratuit des livraisons, afin de mettre fin aux pratiques visant à encourager les achats impulsifs par le consommateur. Pourtant, la livraison a un coût financier et environnemental que le consommateur devrait prendre en compte lors de ses achats. La transparence sur le prix de la livraison doit donc être garantie avant tout achat de biens et de services. Le présent amendement vise à mieux informer le consommateur du prix réel des livraisons effectuées dans le cadre de contrats de vente de biens et de fourniture de services, en prévoyant qu'il s'agit d'une obligation légale précontractuelle pour le vendeur ou le prestataire. Je partage l'objectif de votre amendement, qui permettrait, s'il était adopté, une meilleure information du consommateur. Toutefois, le périmètre de cet amendement touche à un article du code de la consommation qui concerne non pas uniquement les livraisons, mais toutes les prestations non exécutées de façon immédiate.

sans nécessité d'adaptation particulière. Attendre le 1 janvier 2022 ne se justifie donc pas. Avec le présent amendement, nous proposons une application de la mesure à compter de la promulgation de la loi. C'est d'autant plus nécessaire que la crise sanitaire que nous traversons a conduit à une explosion des achats en ligne et à un recours accru à ces pratiques commerciales.

souhaitons donc que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil fixé par décret proposent au consommateur plusieurs options en matière de livraison. Les modalités d'application de cette obligation seraient précisées par décret et sa mise en place est prévue au 1 janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s'y préparer.

décarbonées. La consultation en ligne organisée dans ce cadre avait fait remonter une très forte demande de la part des citoyens : 90 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles souhaitaient avoir davantage de liberté quant aux modalités de livraison, afin de recourir à des solutions plus respectueuses de l'environnement. L'avis est donc favorable.

dont on sait qu'elle est un maillon essentiel, qui, bien optimisé, peut rendre positive la contribution environnementale du e-commerce. Il est également prévu que l'étude confiée à France Stratégie et à France Logistique concernant les plateformes de e-commerce et l'immobilier logistique approfondisse la question des modes rapides de livraison actuellement proposés, qui pourrait constituer l'un des critères permettant de distinguer les plateformes les plus vertueuses. C'est pourquoi il nous semble préférable de mener à bien ces travaux, d'une part, pour objectiver la situation et comprendre quels sont les modes de livraison les plus polluants,

la consultation en ligne réalisée par notre mission d'information a révélé qu'environ 93 % des personnes consultées s'estiment insuffisamment informées des conséquences environnementales de la livraison lorsqu'elles effectuent un achat en ligne. Le présent amendement vise donc à pallier ce défaut d'information, en obligeant les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à un seuil fixé par décret à informer les consommateurs de l'impact environnemental des livraisons des produits qu'elles vendent. Les modalités d'application de cette obligation seraient naturellement précisées par décret ; il pourrait s'agir, dans un premier temps, d'une information délivrée .La mise en place de cette obligation est prévue au 1 janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s'y préparer.

: à chaque fois, il fait démarrer son véhicule, le conduit, puis le stationne à nouveau. Nous sommes en train de pondre une législation dont l'application fera le bonheur des chroniqueurs humoristiques et, pour les plus procéduriers, des avocats sans cause

L'article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités- la LOM -prévoit que les publicités en faveur de véhicules à moteur portent obligatoirement un message faisant la promotion des mobilités actives, telles que la marche ou l'usage du vélo, des mobilités partagées, telles que le covoiturage, ou des transports en commun, de manière à inciter le consommateur au report modal vers des solutions de mobilité moins émettrices de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Dix-huit mois après la promulgation de la LOM, article ne semble toujours pas publié, alors qu'une consultation sur un projet de décret a été engagée il y a tout juste un an. On peut donc s'interroger sur les véritables ambitions du Gouvernement. Notre amendement vise à rappeler la volonté du législateur de voir cette mesure entrer en application sans délai. Quel est l'avis de

faire après cette promulgation ? Tout simplement, les nouvelles normes applicables aux entreprises doivent prévoir un délai d'entrée en vigueur suffisant à compter de la publication du texte. La date proposée du 1 octobre prochain n'est pas réaliste alors qu'on ne connaît pas la date de promulgation du présent du présent texte. Or celui-ci prévoit également de nouvelles obligations d'affichage dans les publicités automobiles. Le Gouvernement souhaite privilégier un cadre stable pour les acteurs économiques, avec une entrée en vigueur simultanée

surtout lorsqu'il s'agit principalement de questions financières, dans le secteur de la publicité comme ailleurs. Nous proposons donc de supprimer un dispositif inopérant, qui renforce les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sans augmenter pour autant ses moyens. C'est par des dispositifs réellement contraignants que nous avancerons sur ces questions, plutôt que par de simples gesticulations.

tout n'est pas encore parfait. Pour ne prendre qu'un exemple, la majorité des enfants et des parents estiment que les bandeaux écrits et non lus sont bien souvent trop discrets, et ce d'autant plus lorsque les publicités exigent de leur part une concentration accrue. Dans un autre domaine, il faut relever le bilan globalement positif des incitations anti-tabac, et ce malgré les pratiques douteuses de certains producteurs qui parasitent les messages inscrits sur les paquets. Ainsi, comme le relève le chercheur Marc Bonhomme dans l'ouvrage collectif,

Par ailleurs, 79 % des fumeurs interrogés pensent qu'ils jouent un rôle d'incitation la discussion ; 68 % d'entre eux estiment que leur présence accroît la réflexion des « accrochés à la cigarette ». C'est bien ce que nous demandons fondamentalement aux politiques sanitaires. Pour citer une nouvelle fois Marc Bonhomme, « il il convient de ne pas trop demander à ces avertissements sanitaires, qui ne constituent qu'une mesure parmi d'autres. Ils favorisent une meilleure responsabilisation de chacun d'entre nous dans notre vie privée. » En gardant tout cela il pourrait être intéressant d'intégrer une dimension environnementale dans les publicités audiovisuelles pour les produits polluants. Alors que le Gouvernement a fait de la réduction de la place de la voiture, ou encore de l'avion, des axes de bataille, inciter leurs utilisateurs à des modes de

traduisant les engagements pris au sein d'un contrat climat conclu entre les médias et les annonceurs, d'une part, et le CSA, d'autre part, afin de réduire la publicité pour les produits polluants. Cette mesure laisse à penser que plus aucune publicité pour les vols long-courriers à destination des collectivités d'outre-mer ne pourra être visible. Alors que les industries touristiques outre-mer, motrices de l'activité locale, sont lourdement et durablement affectées par la crise sanitaire, une telle décision obérerait tout espoir de reprise. Cela fait craindre également que les publicités pour les bananes de Martinique ou de Guadeloupe ne puissent plus être diffusées, l'impact carbone du produit tombant sous le coup du code de bonne conduite défini

peux vous confirmer que les codes de bonne conduite prévus à l'article 5 sont des outils de droit souple ; il serait inopportun de figer dans le texte des dérogations alors qu'aucune interdiction de principe n'est prévue. Il ne semble donc pas nécessaire de préciser dans la loi la prise en compte des spécificités ultramarines. Je tiens

dès 2023. Je suis défavorable à cette disposition, car elle créerait une forte inégalité entre les entreprises de l'audiovisuel public et celles du secteur privé. Surtout, l'objectif de de ce code spécifique me semble déjà en partie satisfait, puisque le code de bonne conduite prévu à l'article 5 permettra de réduire de manière significative les publicités relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement dans l'ensemble des médias audiovisuels, publics comme privés. La mise en oeuvre de ces engagements aura mécaniquement pour conséquence d'augmenter la part de publicités pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement. La mesure proposée est par ailleurs impossible à mettre en oeuvre. Les groupes visés n'auraient pas la capacité de procéder, pour chaque campagne publicitaire, à une analyse concurrentielle sur le caractère substituable des offres de produits et de services moins polluants. Enfin, la suppression de certaines publicités pourrait entraîner des pertes substantielles de recettes pour les sociétés audiovisuelles publiques ; elle risquerait donc de porter atteinte à l'équilibre de leur modèle économique. Or, aux termes de la jurisprudence constitutionnelle et administrative, l'indépendance des médias implique que le législateur garantisse les ressources des sociétés nationales de programme. Aucune compensation financière n'ayant été apportée par le projet de loi, une telle disposition n'apparaît pas conforme à la Constitution.

organise, d'ici au 1 janvier 2024, la suppression des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, suppression applicable à tous les acteurs et non pas seulement aux seules sociétés du service public audiovisuel.

plus de 16 milliards d'euros, dont un tiers se concentrait sur les secteurs de l'automobile, du transport aérien et des énergies fossiles. Or, si une étude de 2013 établissait que 80 % des Français trouvaient la publicité trop intrusive, celle-ci conserve pourtant ses effets d'incitation à l'achat. Au vu de cette situation, l'opposition faite par Aurore Bergé, à l'Assemblée nationale, entre nécessité de lutte contre le dérèglement climatique, d'une part, et relance économique, dont la publicité serait un enjeu central, d'autre part, doit être réinterrogée.

Premièrement, cela contribue une nouvelle fois à creuser le fossé entre secteur privé et service public, et à démunir ce dernier de moyens nécessaires à sa survie et à la qualité de ses programmes. C'est d'autant plus dommageable que les missions du service public audiovisuel mettent l'accent sur la culture et l'éducation et que cela doit englober une sensibilisation accrue des téléspectateurs aux questions climatiques. Deuxièmement, plus grave encore, une telle mesure serait largement insuffisante. Le secteur public ne représente en effet qu'une part minime du marché publicitaire en France. Pour ne prendre qu'un exemple, la fusion voulue entre TF1 et M6 permettrait à ce près de 75 % du marché publicitaire audiovisuel français. Se pose par ailleurs la question des nouveaux secteurs de la publicité, notamment sur internet, qui ne cessent de progresser. Ainsi, la rédaction actuelle de l'article 5 ne permet qu'un progrès très modéré en matière de lutte contre la pollution, tout en précarisant encore un peu plus un service public audiovisuel en difficulté budgétaire, qui doit être au centre de la stratégie de sensibilisation des citoyens.

de la publicité le soir. Elle prévoit qu'un code de bonne conduite conclu avec le CSA organise d'ici au 1 janvier 2023 au plus tard la suppression des communications commerciales sur des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l'environnement sont disponibles. C'est donc une proposition qui rehausse substantiellement l'ambition environnementale du volet relatif à la publicité de ce projet de loi, sans pour autant affecter de façon importante les recettes de nos services publics

laisserait entendre que les médias audiovisuels seraient pleinement en mesure de choisir leurs annonceurs. C'est à mon sens une erreur d'analyse, car les principales responsabilités incombent aux annonceurs et non aux diffuseurs.

de vote. Il est regrettable que ni Mme la rapporteure ni Mme la ministre n'aient répondu concrètement à l'objet des amendements. Madame la rapporteure, si vous considérez qu'il faut absolument maintenir ce à quoi a abouti la commission,

promis depuis trois ans, qui devait tout réorganiser, du financement de l'audiovisuel public à son organisation, sa structuration et sa gouvernance. On en a beaucoup parlé, on nous a beaucoup promis,

En lieu et place de l'interdiction pure et simple de la publicité sur les produits polluants que nous avions proposée dans un précédent amendement, nous avançons ici une autre solution : celle des codes de bonne conduite, dont nous venons de parler.

en matière de publicité alimentaire à destination des enfants s'est révélé peu efficace » et « la France devrait se doter d'une régulation normative de la publicité pour enfant ». Santé publique France a enfoncé le clou à l'été 2020 en relevant que les publicités

quels sont les résultats du refus de légiférer ou de réguler : l'inefficacité est quasi totale. Nous souhaitons ici ne pas reproduire les mêmes erreurs. À défaut, comme nous le proposions à l'article 4, d'interdire directement la publicité pour les produits polluants, nous demandons

Cet amendement est de même nature que le précédent. Il vise à rendre les codes de bonne conduite opposables aux acteurs. Les mauvais résultats constatés dans le dernier « Bilan publicité et environnement » publié en septembre 2020 par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité interpellent. L'Ademe pose clairement la question de la capacité des acteurs de la publicité à réellement se mobiliser pour promouvoir des produits, des services et des imaginaires compatibles avec la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. à prévoir la possibilité pour le CSA de sanctionner les services non vertueux par une mise en demeure et, en cas d'absence de mise en conformité des écrans publicitaires après cette mise en demeure, de prononcer soit une suspension de programme partielle ou totale ou de diffusion publicitaire, soit une sanction pécuniaire, dans les conditions du droit commun des manquements aux obligations des services audiovisuels. Quel est l'avis de la commission

par l'amendement n° 1411, qui vise à renforcer l'effectivité des dispositions de l'article 5 en donnant compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour agir concrètement et orienter la publicité vers des biens ayant un impact moindre sur l'environnement. Je demande donc le retrait de

amendement n'ayant pas été adopté, nous proposons que le CSA engage un processus de consultation et de recherche active

Cet amendement tend à demander au Gouvernement de créer dans le projet de loi de finances pour 2022 une contribution sur les dépenses de communication commerciale des entreprises, en complément de l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants. Les fonds recueillis serviront à promouvoir des messages de sensibilisation à la protection de l'environnement. La publicité, en incitant à la surconsommation une pression quotidienne, a des effets négatifs sur l'environnement, qui sont,, payés par la société et le contribuable. Il est donc normal que ce secteur contribue à compenser ses externalités négatives. Tous les acteurs, y compris économiques, s'accordent sur l'importance de diffuser des messages en faveur de la protection de l'environnement et pour accompagner le changement. Le produit de cette Le produit de cette contribution pourra être utilisé à cette fin. En commission à l'Assemblée nationale, la rapporteure a souligné la santé hétérogène du secteur publicitaire : si la publicité numérique se porte bien, c'est moins le cas de la publicité au cinéma, à la télévision, à la radio et dans la presse quotidienne régionale.

La vidéo est aujourd'hui utilisée de manière intensive. Stockée dans des centres de données, elle est acheminée jusqu'à nos terminaux par les multiples réseaux- câbles, fibres optiques, modems, antennes de réseaux. Tous ces équipements nécessitent de l'électricité, dont la production consomme des ressources et est souvent source d'émissions de CO2. La sensibilisation des consommateurs à l'impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements. Cet amendement vise à fournir une information transparente sur l'impact carbone des consommations de vidéos. Il reprend en partie, d'une part, la rédaction issue des travaux de la commission au Sénat et, d'autre part, l'objet d'un amendement, déposé par notre

les vidéos en ligne représentaient 1 % des émissions de CO2 à l'échelon mondial, soit l'équivalent des émissions de CO2 d'un pays comme l'Espagne en 2018, avant la pandémie.

multiplier les vecteurs législatifs. Avis défavorable.

et la multiplication des nouveaux services proposés aux utilisateurs, lesquels passent désormais des heures sur des applications bien connues à visionner des films, des séries, des documentaires, des clips musicaux ou encore des vidéos postées par des influenceurs. La crise sanitaire a renforcé ces comportements, le visionnage de tels contenus ayant connu une croissance de 35,1 % en 2020. Le présent amendement vise donc à informer le consommateur de l'impact carbone du visionnage de vidéos en ligne lors de leur lecture. L'affichage de la consommation de données et de ses conséquences environnementales constituerait un moyen efficace pour infléchir cette tendance. L'apport de conseils pour réduire cette consommation de données permettrait à ceux qui le souhaitent d'agir en ce sens.

dans le présent article. Cette disposition permettrait une meilleure applicabilité de la mesure au secteur du numérique, ainsi qu'une transparence accrue. En effet, des effets de bord indésirables sont possibles, l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définissant un terminal comme tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations,

sont prévues à l'article 5 , semble pleinement justifiée pour affiner les modèles d'analyse et de suivi développés par des tiers, il convient toutefois d'encadrer cette pratique par un avis du ministre chargé des communications électroniques. Ainsi, l'instauration d'un avis du ministre et de la

6,7 % des émissions de gaz à effet de serre nationales. Cet amendement vise à demander au Gouvernement d'intégrer des objectifs propres au numérique dans la stratégie nationale bas-carbone. Cette stratégie définit un budget carbone correspondant à des plafonds d'émission de gaz à effet de serre, que différents secteurs ne doivent pas dépasser. Elle a donc un rôle structurant dans les politiques publiques mises en place pour atteindre nos objectifs environnementaux.

Cet amendement vise à introduire un budget carbone pour le secteur numérique. La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre associées au numérique est un enjeu essentiel dans la lutte contre le changement climatique. La prochaine stratégie nationale bas-carbone prévoira d'ailleurs des orientations spécifiques au numérique, fondées sur une capitalisation des nombreux travaux en cours sur le sujet. Néanmoins, il faut savoir qu'une partie importante des émissions du secteur numérique ne concerne pas le territoire national, mais a un impact sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions liées à la fabrication des terminaux. En effet, 75 % de l'empreinte carbone du numérique correspond à

et celles dont le maire n'a pas l'intention ou les moyens de le faire. Nous pensons que l'État, garant de l'équilibre des territoires et de l'application des lois, doit conserver sa capacité d'intervention par le biais des préfets concernant les règlements de publicité : c'est ce qu'a permis l'adoption des amendements en commission et nous nous en félicitons

(AMF) n'est d'ailleurs pas favorable à cette disposition. De même, le Conseil d'État la juge inopportune, voire contraire aux objectifs de ce projet de loi, dans la mesure où elle conduirait à fragiliser la protection du cadre de vie de nos concitoyens. nos concitoyens. En outre, le maire engagé dans une réglementation de publicité locale dans le cadre d'un RLP dispose de fait de ce pouvoir de police.

C'est le sens des nombreux amendements identiques que nous avons adoptés en commission.

d'une position d'équilibre satisfaisante, qui permet de décentraliser de manière intelligente sans pour autant créer des risques d'affaiblissement du droit de l'environnement dans les territoires,

à l'échelle de tout un territoire. De même, ce n'est qu'en laissant le pouvoir de police aux préfets que l'on pourra faire en sorte que la réglementation s'applique, non pas de manière aléatoire, mais dans le respect du principe d'égalité sur l'ensemble du territoire national. Chaque maire qui le souhaite doit pouvoir agir pour un meilleur respect du code de l'environnement, mais l'État doit rester le garant du respect du droit et du

restreint très fortement la portée de cette mesure de décentralisation, car la grande majorité des communes sont dépourvues de RLP. En outre, l'article 6 ainsi rédigé complexifie l'exercice de cette police en créant une triple compétence entre le maire,

une telle situation serait source de confusion et pourrait conduire à des dysfonctionnements, les deux autorités compétentes agissant en même temps, de manière désordonnée, ou au contraire comptant l'une sur l'autre pour agir.

destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur la surface, la hauteur, ou le niveau de consommation d'énergie et de nuisance lumineuse du dispositif. Comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis, cet article porterait une atteinte anticonstitutionnelle, car disproportionnée, à la liberté du commerce et au droit de la propriété, en se mêlant de l'aménagement intérieur des magasins, lieux privés, et de la façon dont le commerçant communique auprès de sa clientèle. Il ne tient pas compte de la réglementation existante qui encadre déjà l'extinction et la luminance des enseignes, des publicités et des vitrines, afin de baisser la consommation énergétique et les nuisances lumineuses causées par ces dispositifs.

prévoit que tous les bâtiments tertiaires, dont les bâtiments commerciaux et leurs vitrines, devront réduire leur consommation d'au moins 40 % d'ici à 2040 et de 60 % d'ici à 2060.

L'article 7, tel que modifié au cours de la navette, ne permet pas d'interdire les enseignes et publicités lumineuses derrière les vitrines des commerces ou d'un local commercial : nous nous en sommes assurés dans le cadre de l'examen en commission. Si l'examen à l'Assemblée nationale a permis d'améliorer le dispositif initialement proposé, l'article soumis au Sénat continuait de soulever des difficultés d'ordre économique et environnemental. La commission a donc adopté des amendements identiques, en coordination avec les commissions saisies pour avis, afin de réécrire l'article 7 de manière à répondre

Nous avons notamment sécurisé le dispositif, en limitant au niveau local les possibilités d'encadrement aux seuls horaires d'extinction des vitrines. Je rappelle, par ailleurs, que deux tiers des élus locaux consultés étaient favorables à la régulation prévue dans cet article. J'estime donc que nous avons trouvé un équilibre entre volonté d'encadrement de pratiques

du Gouvernement ? Ces amendements de suppression sont l'occasion d'évoquer les évolutions de l'article 7 adopté par votre commission, laquelle en a profondément modifié le texte. L'article renvoie désormais à un décret en Conseil d'État la fixation des prescriptions en matière d'horaires d'extinction et de consommation énergétique des dispositifs Cette proposition constitue un net recul par rapport à la rédaction issue de l'Assemblée nationale, car elle ne laisse plus aux élus la possibilité d'imposer des prescriptions en matière de surface et de hauteur ; le renvoi à un décret en Conseil d'État ne leur permet plus d'adapter la réglementation nationale aux spécificités de leur territoire. Or l'article 7, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, répondait à un réel besoin exprimé par certaines collectivités qui souhaitent réglementer des enseignes et publicités situées à l'intérieur des vitrines lorsque celles-ci sont destinées à être visibles de l'extérieur. Celles-ci ne peuvent en effet actuellement faire l'objet d'aucune réglementation

L'article 7, tel que le défend le Gouvernement, est donc simplement de bon sens. Je précise, pour M. Demilly, que la version du Gouvernement était validée par le Conseil d'État. Cet article vient combler un vide juridique et donner une compétence supplémentaire aux maires. Nous faisons confiance à ces

Je souhaite donc le maintien de cet article, mais dans une version amendée à l'occasion de la navette, afin de redonner aux élus les leviers nécessaires pour agir. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

est à M. Thomas Dossus. Depuis quelques années, il est désormais possible d'autoriser la pose d'affiches publicitaires gigantesques sur les bâches de chantier, au-delà des seuls monuments historiques. Un nouvel

de ces dispositifs, nous appelons à raison garder et à diminuer de manière draconienne leur taille pour les réduire à douze mètres carrés au maximum, comme c'est actuellement le cas pour les panneaux publicitaires ailleurs en ville et sur tout le territoire. Cet amendement a ainsi pour objet de réduire la pollution visuelle, de nous mettre davantage en cohérence avec le reste du code de l'environnement et de freiner les appels à la surconsommation. Quel

est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Diminuer la surface occupée par les affichages publicitaires dans l'espace public répond effectivement à la demande de la Convention citoyenne pour le climat. C'est pourquoi le ministère de la transition écologique porte un projet de décret qui va modifier le code de l'environnement, notamment pour réduire de douze à dix mètres carrés et demi la surface unitaire maximale des publicités et des enseignes, qu'il s'agisse de dispositifs installés sur les murs, scellés au sol ou installés directement sur le sol.

avec leurs compétences, le dérèglement climatique. Nous connaissons désormais les effets néfastes de la publicité sur le climat, ses appels à la surconsommation participant à l'épuisement des ressources et à la pollution de l'environnement. Il n'est plus possible de laisser librement devant nos yeux, sans réaction des autorités, des publicités pour des SUV, des smartphones ou des compagnies aériennes. Aujourd'hui, au coeur des villes, des publicités géantes affichent des produits et des services concourant directement à la dégradation du climat, sans que les maires et les présidents d'EPCI aient leur mot à dire, en contradiction totale avec leurs efforts menés par ailleurs. menés par ailleurs. La lutte contre les dérèglements climatiques doit être globale et s'appuyer sur tous les acteurs du territoire, au premier rang desquels les édiles. Si ceux-ci peuvent travailler sur plusieurs éléments, comme la taille des dispositifs publicitaires ou la densité de l'emplacement, ils ne peuvent agir sur leur contenu ; si ces bâches participent parfois de la rénovation thermique des bâtiments dans une optique de baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale, le contenu même de certaines de ces publicités a pour conséquence une forte hausse des émissions. Face à ce paradoxe, les maires et les présidents d'EPCI doivent être accompagnés pour asseoir une politique cohérente dans leur lutte locale contre le dérèglement climatique

La question de la pollution lumineuse est malheureusement absente du présent projet de loi. Pourtant, ses ravages sur la biodiversité ne sont plus à démontrer : perturbation du cycle de vie naturel des animaux, conséquences sanitaires sur l'homme, impact sur l'observation du ciel nocturne, consommation d'énergie accrue. Tous ces effets sont bien documentés et devraient être faire de l'attention du législateur. Cet amendement vise à réparer cet oubli. Depuis la loi Grenelle II, les maires sont dotés de compétences de régulation des sources lumineuses sur leur territoire. sont particulièrement chargés de contrôler le respect de la loi, et de s'assurer que les installations lumineuses privées installées sur leur commune se plient aux prescriptions des textes en vigueur. Or, pour y parvenir, ils ne disposent que d'un simple pouvoir de mise en demeure. Nous souhaitons leur confier un pouvoir d'ordonner proportionnée au niveau des nuisances produites. Une amende journalière paraît être un outil efficace pour s'assurer du respect de la loi. Nous proposons également que soit clairement fait mention dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) de la nécessaire maîtrise de l'éclairage dans l'espace public et de la lutte contre les nuisances lumineuses.

En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d'environ 5 térawattheures par an, soit 1 % de la consommation électrique nationale, la part de l'éclairage public dans l'empreinte écologique de notre pays est loin d'être négligeable. Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd'hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser des économies rapides et importantes sur leurs factures d'énergie et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d'entretien, si des automatismes intelligents d'allumage et d'extinction sont associés au remplacement des luminaires. Pour accélérer le renouvellement des réseaux d'éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls EPCI compétents en matière d'éclairage public l'obligation de prévoir, dans le programme d'actions défini dans le PCAET qu'ils sont tenus d'adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d'énergie de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses. Le présent amendement a donc pour objet d'étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l'article L. 2224-37-1 du code ce qui n'emporte aucune augmentation de charge pour le bloc communal -, qui peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l'élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d'éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.

qu'un, deux, voire trois immeubles sont continuellement recouverts de bâches de plusieurs centaines de mètres carrés. Nous vous proposons donc de revenir à une logique de mécénat pour les entreprises qui souhaitent financer la restauration du patrimoine

J'admets que ce dispositif n'est pas très satisfaisant, mais il permet de dégager des fonds pour la restauration des monuments historiques et de consacrer ainsi une plus grande part du budget de l'État à d'autres monuments dont la situation ne permet pas qu'ils en bénéficient,

Contrairement à ce qu'indique l'objet de l'amendement, l'article 8, tel que modifié par la commission, n'interdit pas les publicités dans les airs. Nous sommes en effet revenus à la rédaction initiale du projet de loi, qui se contentait de créer un régime de sanction associé à la régulation de la publicité dans les espaces naturels. Je rappelle que l'exécutif dispose déjà de la possibilité d'interdire la publicité dans les airs par voie réglementaire. L'avis est donc défavorable.

modes polluants de publicité : les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.

un catamaran déploie un panneau numérique géant de trente-deux mètres carrés visible depuis les plages de Cannes par les baigneurs. Ce sont là deux exemples d'un avenir auquel personne n'aspire, un avenir dans lequel la technologie est poussée jusqu'à l'absurde pour accélérer l'invasion complète et totale de l'environnement public par les injonctions publicitaires, à l'aide de dispositifs de plus en plus énergivores. Le législateur ne doit pas être réduit à réagir avec un train de retard lorsque la situation est déjà mal engagée. Nous pouvons parfois prendre les devants, identifier les sujets qui pourraient poser problème à l'avenir et les traiter avant que le problème ne

Cet amendement vise à rétablir l'inscription dans la loi de l'interdiction de la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef. Cette insertion au niveau législatif, souhaitée par les députés, garantit une meilleure lisibilité du dispositif, ainsi que son effectivité. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite assurer la préservation globale des plages, qui doivent rester des milieux naturels protégés de toute pollution visuelle. Dès lors, le présent amendement vise à pallier le vide juridique existant, s'agissant de la publicité diffusée au moyen d'embarcations exploitées à des fins publicitaires sur les mers territoriales. Comme vous, en effet, je suis choquée : on ne ferme pas la porte à une forme de publicité pour qu'elle rentre par la fenêtre. On n'interdit pas la par avion sur les plages pour qu'elle revienne par bateau. Il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Je propose donc d'interdire la pratique qui consiste à mettre des écrans publicitaires géants sur des bateaux. Les vacanciers ont droit à un peu de tranquillité. Le Gouvernement a en outre conscience de l'importance de ne pas déstabiliser le secteur des événements sportifs. C'est pourquoi le présent amendement vise de manière ciblée l'interdiction de la publicité diffusée par embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires. Cette rédaction exclut donc notamment du périmètre de l'interdiction les navires qui sont utilisés pour les événements sportifs nautiques. Le

qui ne vise que l'activité de tractage de banderoles, nous paraît équilibrée. Il est cependant proposé de reporter l'entrée en vigueur au 1 janvier 2023, afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques, notamment les très petites entreprises, qui seront touchés. Quel est l'avis de Il ne nous semble pas opportun d'inscrire dans la loi l'interdiction des avions publicitaires ou de la publicité des véhicules terrestres, à moteur ou des embarcations à moteur. Des interdictions peuvent déjà être décidées par le Gouvernement, par voie réglementaire, sur le fondement de l'article L. 581-15 du code de l'environnement. Pourquoi donc rendre la loi bavarde et légiférer pour encadrer des pratiques qui peuvent déjà l'être ? J'ajoute que des interdictions par voie réglementaire seraient sans doute plus précises

hormis les cas où une étiquette autorisant cette distribution est apposée sur la boîte, remplaçant ainsi le principe du Stop Pub par celui du Oui Pub.

Pourtant, mes chers collègues, chaque année, près de 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres. Cela représente 800 000 tonnes de papier, soit 30 kilogrammes par foyer en moyenne. La distribution de prospectus publicitaires est un non-sens écologique. La fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie ; elle favorise la déforestation. Au surplus, les prospectus publicitaires étant lus par moins de 15 % des destinataires, cette méthode semble inopérante d'un point de vue commercial. Certes, Certes, la loi AGEC a apporté des avancées en la matière, avec l'expérimentation du dispositif Stop Pub. Mais si les citoyens souhaitent aller plus loin que ces dispositions, quel est le problème ?

allons plus vite, et augmentons les pensions : ce sera socialement plus juste ! Nous estimons, pour conclure, qu'il est temps d'en finir avec ce gaspillage, et qu'il convient de passer au Oui Pub, laissant à chacun la liberté, et je dirais même la responsabilité, d'affirmer sa disponibilité pour ce type de démarchage.

C'est un gâchis invraisemblable, qui frise l'indécence. Combien d'arbres abattus, combien de processus de recyclage inutiles mis en oeuvre ? Combien de déchetteries encombrées, combien de véhicules, de moyens logistiques polluants déployés, le tout pour distribuer des documents qui ne seront pas lus

d'imprimés publicitaires sans adresse qui ont été distribués, soit 30 kilogrammes par foyer et par an, souvent jetés sans même avoir été lus. Le bilan s'élève à 736 000 tonnes de CO2. L'objectif de cet article est de lutter contre ce gaspillage. une enquête de l'Ademe indique que 70 % des répondants se déclarent « très » ou « plutôt ouverts » à ce qu'un système inverse au Stop Pub soit testé et appliqué dans leur commune. Je comprends le souhait

de prospectus publicitaires non adressés, sauf demande des habitants sur la boîte aux lettres. Cet article ne vise ni la distribution de prospectus dans la rue ou dans les centres commerciaux ni la publicité adressée. Par ailleurs, d'autres canaux pour faire de la publicité existent, en dehors de la distribution de documents et du canal numérique, comme les affiches, la publicité orale dans la rue, etc. Les emplois correspondant à la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres pourront être redéployés vers ces canaux. De plus, pour ce qui est de l'emploi, ce sont la conception et l'impression du premier exemplaire qui requièrent de la main-d'oeuvre.

personnes peuvent avoir envie ou pas de s'afficher « écolo ». Pourquoi alors privilégier le gaspillage par défaut plutôt que la prévention du déchet ? L'autocollant Oui Pub peut être conçu aussi de manière très discrète, dès lors qu'il est connu du distributeur. Il peut s'appeler, par exemple,

Des études convergentes mettent en évidence l'impact environnemental significatif de la publicité par voie numérique. Le groupe La Poste, par exemple, a publié, le 15 octobre dernier, une étude comparative de l'impact environnemental des communications papier et numérique. Le but de cette analyse était de comparer l'impact environnemental des supports de la relation client- mailing, flyer, facture ... -dans leur version papier et dans leur version numérique, selon seize indicateurs répartis en cinq catégories l'impact sur les écosystèmes, les ressources, la santé humaine, l'utilisation de l'eau et le changement climatique. Les résultats révèlent que le papier est plus favorable en moyenne que le numérique pour treize indicateurs environnementaux sur Le marché de la publicité sur internet représente aujourd'hui 6 milliards d'euros, soit 40 % du total des dépenses publicitaires. Ces données en font aujourd'hui un vecteur de publicité majeur et une source de consommation d'énergie importante. Notre amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 1 janvier 2023, un rapport sur l'impact environnemental des campagnes publicitaires effectuées par voie numérique. Celui-ci permettra de mettre en place une trajectoire pour assurer la neutralité carbone d'ici à 2050 du secteur de la publicité sur internet. Nous le cas échéant des mesures de régulation. Le principe que vous défendez, monsieur le sénateur, était inscrit dans la rédaction qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. J'y suis donc plutôt favorable, mais la rédaction de votre amendement pose un certain nombre de problèmes que je n'ai pas pu expertiser.

se référer plutôt à un « accord » du consommateur. En effet, en pratique, il est peu vraisemblable que le consommateur réclame un échantillon. Dans le cadre d'une relation commerciale, c'est le professionnel qui propose et le client qui accepte. Si certaines bonnes pratiques consistent à proposer un échantillon au consommateur et à le lui remettre en cas d'accord, celles-ci restent volontaires et non généralisées. Rendre une telle obligation contraignante en l'inscrivant dans la loi représenterait une amélioration par rapport à la situation actuelle.

Gouvernement ? Ces amendements ont pour objet d'interdire la fourniture d'échantillons d'un produit à un consommateur sans son « accord », alors que la rédaction actuelle fait référence à une « demande » de sa part.

tant pour le professionnel que pour le consommateur. Ainsi, il me semble souhaitable de maintenir la rédaction actuelle d'interdiction de remise d'échantillons sans demande de la part du consommateur. C'est pourquoi je souhaite le retrait de ces amendements, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable. Madame Dumas, l'amendement

ou d'abonnement à une publication de presse comme suffisant pour que celle-ci emporte « présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir » reviendrait à supprimer toute possibilité d'intégration d'échantillon dans les publications. Or l'intégration d'échantillons dans les publications de presse fait partie intégrante du modèle économique d'un grand nombre d'entre elles. Dans un contexte où les revenus publicitaires de la presse magazine sont déjà fragilisés, cette mesure risque d'affaiblir encore le secteur. En outre, sans l'avantage concurrentiel majeur que constituent les échantillons par rapport aux autres médias, celle-ci ne ferait qu'accélérer le transfert des recettes publicitaires vers le digital, et renforcerait le déséquilibre en faveur des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). La suppression de l'exemption pour les échantillons presse serait donc véritablement punitive pour le secteur de la presse, alors même que les entreprises cosmétiques, particulièrement concernées, font des efforts pour une meilleure écoconception des échantillons, en rationalisant leur format et en améliorant la recyclabilité de leurs emballages.

de la commission ? La commission a adopté un amendement qui supprime l'exception accordée à la presse papier concernant l'encadrement de la distribution des échantillons. Les auteurs de cet amendement avaient considéré que cette exception risquait de créer une forte augmentation du nombre d'échantillons

de fourniture d'un échantillon auprès d'un éditeur de presse, qu'il s'agisse de l'achat d'un journal ou d'un magazine. L'interdiction de fourniture d'échantillons aurait des conséquences importantes sur le modèle économique de la presse magazine, dans un contexte où les revenus publicitaires de la presse sont déjà très fragilisés, avec une baisse de 52 % du chiffre d'affaires publicitaire entre 2009 et 2019, suivie d'une chute de plus de 30 % de ce chiffre d'affaires, en 2020. J'entends les craintes qui ont été exprimées en commission quant à une augmentation du nombre d'échantillons dans la presse papier.

En droit français, il existe un flou juridique sur cette définition. D'une part, l'échantillon est désigné comme un « avantage de valeur négligeable » dans le code de la santé publique ; d'autre part, en droit de la consommation, on s'y réfère comme à un produit « d'une valeur maximale

Autre illustration, ce flou juridique pose la question de la dégustation de produits alimentaires proposée dans certains commerces. Il s'agit de savoir si les produits distribués aux consommateurs sont assimilables ou non à des échantillons.

puisque le décret encadrera les conditions et donc le périmètre d'application précis de cet article.

de l'emballage et de la formule, l'impact de la fabrication du produit, le transport des matières premières qui compte pour deux tiers de la note. Les six autres critères portent sur l'impact sociétal, s'agisse de la localisation en France de la production, de la labellisation bio, du commerce équitable, ou de la certification Origine France Garantie. L'engagement sociétal est un élément particulièrement important pour ce groupe qui- il faut le rappeler -est contrôlé par une fondation.

Afin de renforcer son attractivité et de s'assurer que la filière participe clairement au développement du pouvoir d'achat des consommatrices et des consommateurs, nous proposons d'agir sur le taux de TVA qui s'applique aux produits non emballés, en libre-service, dans les grandes surfaces. amendement prévoit donc d'exonérer les produits alimentaires vendus en vrac, aujourd'hui taxés au taux de 5,5 %. Une telle disposition semble juste et souhaitable, lorsque l'on sait que la vente directe des agriculteurs aux consommateurs est exonérée exonérée de TVA. Nous proposons parallèlement de fixer le taux de TVA des produits non alimentaires à 10 % au lieu de 20 %. Il s'agit d'un exemple concret permettant de conjuguer l'exigence d'un renforcement du pouvoir d'achat de nos concitoyens et la nécessaire transition écologique, dans la logique de la lettre de mission de la Convention citoyenne. Nous espérons donc que cet amendement sera enfin adopté. Cet amendement vise à encourager le développement de la vente en vrac, dans l'esprit des dispositions de l'article 11 du présent projet de loi. Il prévoit d'appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumises. L'objectif est d'inciter à l'achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et, plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source. L'avis est défavorable sur les deux amendements, mais pas pour les mêmes raisons. En ce qui concerne l'amendement n° 153, si la directive de 2006 autorise la mise en place de taux réduits pour l'alimentation, il n'est en revanche pas possible d'exonérer complètement de TVA ces produits. vous comprendrez donc pourquoi l'avis est défavorable. Quant à l'amendement n° 1625, le principe de neutralité de la TVA interdit d'appliquer des taux différents à un même produit selon le procédé de fabrication ou de distribution. Le droit de l'Union européenne détermine de manière très limitative les livraisons de biens et des prestations de

ce travail a été mené conjointement avec la commission des affaires économiques. Nous avons clarifié le texte pour rendre l'obligation prévue à l'article 11

25 % de la surface des magasins à l'horizon 2023 et 50 % à l'horizon 2030, le tout pour les commerces de plus de 300 mètres

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas l'adoption d'une mesure qui pourrait favoriser la grande distribution au détriment des plus petits commerces. Aussi, comme la Convention citoyenne pour le climat, nous proposons la mise en place de la vente en vrac dans tous les magasins de vente au détail : le seuil de 20 % fixé à l'horizon 2030 nous paraît à la fois opportun et tout à fait raisonnable. On le sait, nos concitoyennes et nos concitoyens plébiscitent la vente en vrac, mais beaucoup d'entre eux sont freinés par l'absence de telles surfaces de vente dans leurs magasins. Tel est l'objet de notre amendement.

présent amendement tend à garantir la diversification des produits vendus sans emballage primaire dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 11. Je partage le diagnostic selon lequel l'objectif visé n'apportera pas une réponse homogène selon les produits ou les réseaux de vente Le Gouvernement est bien conscient que la vente en vrac, et plus généralement la vente sans emballage primaire, est aujourd'hui mûre dans certains secteurs, comme celui des fruits et légumes, des produits frais à la coupe ou des produits secs, mais qu'il reste des solutions techniques à trouver pour l'étendre

Dans une logique de réduction de l'empreinte carbone des produits proposés à la consommation, de soutenabilité et de développement d'une consommation locale et de valorisation du patrimoine alimentaire local, cet amendement de Victorin Lurel vise à mettre en avant, dans les surfaces de vente, les produits issus de la production locale lorsque cela est possible ou, le cas échéant, les produits provenant de l'aire géographique où se situe

Cabanel, pour présenter l'amendement n° 221 rectifié. L'article 11 vise à accélérer la vente en vrac dans les moyennes et grandes surfaces. Si la réduction des déchets issus d'emballages ménagers est un objectif que nous partageons tous, la généralisation de la vente en vrac est une solution particulièrement contre-productive pour la filière viticole. L'utilisation du verre est fondamentale pour le conditionnement du vin. Participant de l'identité du vin, la bouteille est le contenant historique, traditionnel et le mieux adapté à son vieillissement.

Enfin, la bouteille en verre est de plus en plus souvent le support d'informations obligatoires, telles que les identifiants de traçabilité, le numéro du lot et, bien sûr, l'étiquetage qui offre de précieux renseignements aux consommateurs.

vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles, voire pas compatibles du tout, avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402, 403, 438 et 520 A du code général des impôts relatifs

n'envisage de vendre du champagne en vrac